», pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau inscrits dans le dispositif de double projet du pacte de performance, grâce au mécénat. Cette mesure est d'autant plus importante que nous accueillerons bientôt les jeux Olympiques.

malgré les mesures d'urgence, les secteurs du spectacle vivant, du cinéma et du livre, ainsi que les musées, sont confrontés à une perte de recettes sans précédent, avec des perspectives de reprise incertaines. Parallèlement, la paralysie de l'économie incite peu les entreprises et les particuliers à investir le dispositif fiscal associé aux opérations de mécénat. Pourtant, le premier confinement a donné lieu à un élan de solidarité, qu'il importe de prolonger en renforçant l'attractivité du mécénat. C'est pourquoi il est proposé d'augmenter, à titre exceptionnel- j'y insiste -, le taux de réduction fiscale de 60 % à 80 % pour les montants inférieurs à 2 millions d'euros et de 40 % à 60 % pour les montants supérieurs. L'amendement

parole est à Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à lutter contre les écarts excessifs de revenu au sein de l'entreprise, en s'appuyant sur l'outil fiscal. Depuis deux décennies, nous assistons à l'explosion des écarts de rémunération au sein des entreprises. Ces injustices salariales nuisent grandement à la performance des entreprises et fragilisent la cohésion sociale. Puisque nous sommes dans l'incapacité constitutionnelle de limiter à la source ces écarts de rémunération, nous défendons l'idée d'une régulation fiscale au sein de l'entreprise : au-delà de douze fois le salaire minimal, les charges salariales ne seraient plus déductibles du calcul de l'impôt sur les sociétés.

Cette mesure me paraît particulièrement pertinente au coeur de la crise de la covid-19, alors que l'État a besoin de ressources nouvelles et justes pour limiter la dette publique. En luttant contre les inégalités, notre pays peut renouer avec un esprit de solidarité et d'entreprise l'avis de la commission ?

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement vise à favoriser les commerces de centre-ville et de centre-bourg, particulièrement touchés par la crise face à la concurrence déloyale des grandes surfaces commerciales, qui sont implantées le plus souvent en zone périurbaine et qui concourent à l'artificialisation

est d'ailleurs la conclusion du rapport n° 19-100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux à la demande du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, rapport dont cette proposition s'inspire largement. L'Assemblée nationale a prévu la prorogation du dispositif pour deux ans, mais celui-ci mérite d'être largement amélioré. En outre, cette simple prorogation n'offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques, car les questions forestières se traitent sur le temps long. Cet amendement vise donc à améliorer la lisibilité du dispositif et à le rendre plus stable. En ce qui concerne le DEFI acquisition, il est proposé de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l'unité de gestion grâce à l'acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n'incite pas les personnes possédant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à

de supprimer l'obligation de conservation des parts de groupement forestier ou de forêt ; d'augmenter la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire, et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier d'augmenter le taux du crédit d'impôt à un taux ordinaire de 30 %, y compris pour le DEFI contrat, et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.

que ce dispositif est le plus intéressant pour eux. Il est vraiment nécessaire d'y apporter les améliorations pointées dans le rapport d'avril 2020.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à prolonger jusqu'en 2024 le crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers et à supprimer un seuil réglementaire. Le crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers permet d'entretenir et de régénérer la forêt, ce puits de carbone indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques.

ou intégrer un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, ce critère étant pénalisant pour les petits propriétaires, qui sont aussi des acteurs essentiels de la biodiversité. En effet, l'adhésion à une organisation de producteurs ou l'intégration dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier impose des contraintes difficilement compatibles avec des petites surfaces et pénalisantes vis-à-vis des entreprises forestières indépendantes.

n° II-1447 rectifié. L'article 199 B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements qu'ils réalisent outre-mer. Les investissements supérieurs à 250 000 euros peuvent être réalisés au moyen d'une société par actions- société anonyme, ou SA, ou d'une société par actions simplifiée, ou SAS -, mais ce n'est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros qui ne peuvent être effectués qu'au moyen d'une société de personnes, une société en nom collectif, ou SNC, dans la plupart des cas. termes de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l'objet d'une offre au public ou d'un placement privé, en particulier les actions émises par les SA ou SAS. Par conséquent, la distribution des opérations d'investissement outre-mer, les parts de SNC qui ne sont pas des titres financiers ne peuvent pas faire l'objet d'une offre au public ou d'un placement privé. La modification proposée, qui permet le recours aux sociétés par actions- SA ou SAS -pour tous les investissements réalisés outre-mer, quel que soit le montant investi, sécuriserait juridiquement les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français, tout en leur assurant une meilleure protection. la distribution des titres financiers relevant de la directive européenne Mifid II vise à renforcer la protection des investisseurs à l'égard des institutions financières en exigeant de leur part des informations claires et non trompeuses. De plus, les associés d'une société en nom collectif sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société, ce qui n'est pas le cas pour les actionnaires d'une société par actions qui ne sont responsables qu'à hauteur du capital qu'ils détiennent dans la société. Enfin, le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, s'exerce sur les acteurs du montage et de la distribution des titres financiers, ce qui n'est pas le cas pour les parts de SNC qui sont des « biens divers proposée permettra enfin de mettre un terme à une contradiction manifeste entre le code général des impôts, qui autorise la commercialisation des programmes d'investissement outre-mer sous forme de SNC, et le code monétaire et financier, qui l'interdit.

mesure permettrait de répondre pour partie aux besoins en logements sociaux à La Réunion, en particulier en matière de logements étudiants. Forte d'une démographie étudiante en croissance régulière, La Réunion présente un manque de logements étudiants, ce qui constitue un frein à l'attractivité de l'université de ce territoire. Contrairement à la situation dans les autres DROM, le quota actuel est systématiquement saturé à La Réunion depuis plusieurs années, entraînant la mise en échec de nombreuses opérations et l'augmentation des demandes insatisfaites pour ce type de logements. Quel est l'avis de la commission ?

néanmoins que la limitation du nombre de PLS éligibles permet de garantir la vocation première de l'article 244 X du code général des impôts, à

de sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs. employeurs. Cette extension ne concerne que les régimes légalement obligatoires, mais institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis. Elle ne vise donc en réalité que l'Agirc-Arrco, régime complémentaire de droit commun pour les salariés du secteur privé. De ce fait, certains employeurs de salariés affiliés à des régimes obligatoires institués par la loi, qui ne peuvent pas bénéficier de l'extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire prévue par le code en vigueur, pourraient se retrouver privés du bénéfice de la compensation du CICE pour une partie de leurs salariés. Cette situation ne concerne que les employeurs des salariés affiliés

monsieur Lurel,

les reliquats sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires. Ce n'est que dans un second temps, s'il y a des besoins de financement pour les transports, qu'on

Afin d'encadrer l'extinction de ce dispositif, ces derniers pouvaient continuer à titre transitoire d'en bénéficier, sous réserve que les investissements engagés avant le 31 décembre 2018 aient été achevés au plus tard le 31 décembre 2020. Cela étant, en raison du contexte pandémique, les chantiers ont été interrompus lors du premier confinement, et les travaux engagés n'ont pu être achevés dans les temps impartis. Aussi, cet amendement a pour objet de proposer la prorogation du bénéfice du CIIC, pour les meublés de tourisme, d'une année supplémentaire pour les projets engagés avant le 31 décembre 2018. Cette disposition permettrait notamment aux entreprises locales d'assurer la fin des chantiers en cours sans avoir à craindre des actions judiciaires de la part des acquéreurs privés pour non-livraison dans les temps impartis.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers non-résidents d'une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux interne de 30 %. La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent de 10 % ou 15 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés. L'arbitrage de dividendes permet d'échapper à cette retenue à la source, c'est-à-dire à l'impôt, grâce à deux types de montages un montage interne, substituant temporairement au non-résident un résident français, qui est souvent une banque, et un montage externe, qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables. Cet amendement vise à faire échec à ces manipulations.

Cette mesure ne coûtera pas grand-chose à l'État, parce que nous pensons très sincèrement que la croissance des PME suscitera une recette fiscale qui compensera très largement les pertes de l'État. J'ajoute enfin

Vous proposez de transposer le dispositif ISF-PME à l'impôt sur la fortune immobilière pour soutenir le développement des petites entreprises. Cependant, l'impôt sur la fortune immobilière ne vise à taxer que les seules capacités contributives résultant de la détention directe ou indirecte d'un patrimoine immobilier

monsieur le ministre,

Cette niche fiscale n'a produit que 322 millions d'euros d'investissement cette année, ce qui représente 0,26 % du montant des prêts garantis par l'État consentis pendant cette pandémie. On voit bien qu'on est loin du compte en matière de financement des entreprises.

Madelin. Cet amendement, qui me semble répondre à un certain nombre de critères d'alerte évoqués de part et d'autre, a pour objet de proroger d'une année le dispositif Madelin amélioré,

Les fonds propres des PME sont mis à mal par la crise sanitaire. Même si cela ne permettrait d'engranger que quelques centaines de millions d'euros, c'est un long chemin que de faire des Français des actionnaires. Cela n'est pas dans notre culture, mais nous y arriverons.

la réduction d'impôt au titre de l'investissement en fonds propres réalisé par les personnes physiques au sein des entreprises dites « foncières solidaires », qui bénéficient de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ». En effet, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs modifications ces dernières années : la majoration du taux de réduction d'impôt est passée de 18 % à 25 % en 2018, mais le décret n'a été publié que le 7 août

Je vous remercie

chaque année pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce plafonnement global s'applique à la quasi-totalité des dispositifs fiscaux accordés, tels que l'IR-PME, l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants ou encore les dépenses engagées pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. Il ne s'applique toutefois pas aux dons. Toujours dans la logique visant à mobiliser l'épargne des citoyens vers des projets à fort impact social et environnemental par le biais d'investissements au capital d'entreprises solidaires, il nous semble que l'application d'un plafond plus élevé pour les investissements solidaires serait une bonne mesure incitative. En effet, les citoyens auraient ainsi une marge plus importante pour investir dans les entreprises solidaires, sans que cela oblige ces dernières à renoncer à d'autres crédits d'impôt importants. À l'instar de la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer ou des souscriptions au capital d'une société de financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les réductions d'impôt accordées pour les investissements directs en fonds propres au capital d'une entreprise solidaire

à Mme Isabelle Briquet. Les entreprises solidaires ayant pour objet d'agir sur la transition énergétique se développent et contribuent à amplifier les initiatives citoyennes pour lutter contre le changement climatique. Contrairement aux acteurs traditionnels du marché de l'énergie, ces entreprises solidaires fonctionnent selon un modèle économique particulier et s'appliquent un principe de lucrativité limitée. Elles oeuvrent dans un secteur de l'énergie à forte intensité capitalistique et, du fait de leur modèle, font face à un risque plus élevé. Cet amendement, suggéré par Finansol, vise à soutenir les entreprises actives dans les ENR citoyennes, en leur permettant de bénéficier du dispositif d'incitation à l'actionnariat solidaire sociale, dispositif dont elles sont aujourd'hui exclues lorsqu'elles exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif de rachat de la production d'électricité renouvelable ou d'un contrat de complément de rémunération. Nous pensons que le soutien de la puissance publique pour orienter l'épargne privée vers ces projets et faciliter ainsi les levées de fonds des entreprises actives dans les ENR citoyennes serait opportun. Quel est l'avis de la commission

Je persévère ! Aujourd'hui, le taux d'enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par l'article 726 du code général des impôts.

afin que ces dernières puissent bénéficier du même taux que celui qui s'applique aux titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Quel est l'avis de la commission

En effet, le taux dérogatoire constitue une aide d'État, qui devra être décomptée du plafond des versements éligibles à cette réduction d'impôt, de manière à respecter les règles européennes en la matière. Il y a donc un risque d'effet contre-productif. Deuxièmement, sur le plan constitutionnel, il m'apparaît difficile de créer une inégalité de traitement entre les personnes morales à prépondérance immobilière, selon

le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà. Nous ne sommes pas favorables à l'abandon de la condition d'exclusivité géographique du fonds d'investissement de proximité outre-mer, dans un double souci d'alignement

à s'inscrire dans le prolongement des recommandations de la commission d'enquête du Sénat constituée à la suite de l'accident industriel de Lubrizol et Normandie Logistique, à Rouen, le 26 septembre 2019, et à améliorer l'efficacité de la politique de prévention des risques industriels et technologiques. En l'espèce, il s'agit de mieux coordonner le crédit d'impôt prévu à l'article 200 A du code général des impôts et le dispositif de financement prévu à l'article L. 515-19 du code de l'environnement, qui permet de soutenir les propriétaires de logements inclus dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques pour la réalisation des diagnostics et travaux sur leur logement, quand ces travaux sont rendus nécessaires par les prescriptions dudit PPRT. Surtout, le II de l'amendement permettra de traiter le cas des 1 500 ménages qui ne pourraient plus bénéficier d'un financement de la part de l'exploitant industriel à l'origine du risque et de la part des collectivités territoriales, et ce à compter du 1 janvier 2021, conformément aux échéances fixées par l'article L. 515-19 du code de l'environnement. Ce financement représente une prise en charge conséquente pour les propriétaires concernés, à hauteur de 50 % des dépenses nécessaires, dans la limite de 10 000 euros par logement. Je remercie le Gouvernement d'avoir lui aussi déposé un amendement sur ce sujet important. Un an après l'accident majeur de Rouen, nous devons collectivement être à la hauteur des enjeux. La parole

Acheter un bien immobilier ou un terrain devient pratiquement impossible pour un insulaire, sachant qu'un Corse sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Cette situation crée une fracture sociale et territoriale forte, que nous proposons de réduire en créant une taxe spécifique sur les résidences secondaires sur l'ensemble du territoire de l'île, perçue par la collectivité de Corse, afin d'alimenter, notamment, les moyens nécessaires à l'exercice du droit de préemption, qu'il faut par ailleurs renforcer. Préférentiellement, pour des raisons éthiques, morales, sociales et culturelles, la notion jurisprudentielle de centre des intérêts matériels et moraux pourrait être adaptée au cas de la Corse, afin de ne pas pénaliser les propriétaires de résidences secondaires dans l'intérieur de l'île. Le principe serait de fiscaliser l'ensemble des résidences secondaires de l'île, quelle que soit l'origine du propriétaire, à la condition de permettre à la collectivité de Corse de fixer les taux et assiette, mais surtout de lui donner la capacité de différencier les taux selon les communes, à partir de critères objectifs- objectifs- évolution du prix du foncier ou du taux de croissance des bases locatives, densité démographique, taux de résidences secondaires, etc. -, et en y intégrant des possibilités d'exonération selon les barèmes de revenus, à définir sur critères sociaux. Quel

très important pour les communes d'Île-de-France. À mon avis, il pose aussi la question de la transparence de l'information donnée aux parlementaires au moment de de la relation de confiance dans la discussion budgétaire, notamment en cette période de crise, où les augmentations de dépenses et les pertes de recettes atteignent des

Les montants seront importants, aussi, pour d'autres collectivités d'Île-de-France. Qu'il faille des moyens pour l'Afitf, c'est évident. Qu'il faille préserver les ressources d'Île-de-France Mobilités, nous le disons tous sur ces travées, et nous avons d'ailleurs dû nous battre pour cela dans le cadre du PLFR 4.

d'une disposition surprise au PLFR 4, sur laquelle nous ne pouvons en aucun cas revenir dans le PLF pour

notre ligne directrice. Enfin, gardons à l'esprit que la fiscalité dérogatoire de l'épargne logement n'est peut-être plus si justifiée que par le passé, en raison notamment de la forte baisse des taux d'intérêt.

répartition des amendes de stationnement au titre de 2021

présenté par Mme Paoli-Gagin,

pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Dès lors que l'affectation agricole du bâtiment est établie, le fait qu'il appartienne à un exploitant isolé ou à une société exclusivement constituée

En effet, les personnes de conditions modestes pouvaient bénéficier jusqu'alors de plusieurs dispositifs d'allégements, qui donnaient lieu, eux-mêmes, au versement d'une compensation aux collectivités locales. En 2019, les communes ont ainsi perçu 1,3 milliard d'euros de compensations d'exonération de taxe d'habitation au titre des allégements en faveur des ménages modestes et les établissements

de recettes équivalentes à l'ancienne taxe d'habitation au titre des logements sociaux qui seront construits à l'avenir. Or la construction de logements sociaux entraîne déjà d'importantes pertes de recettes fiscales pour les communes et les EPCI. En effet, elle ouvre droit à une exonération de taxe foncière au bénéfice des bailleurs pour une durée allant de quinze à trente ans. Les compensations versées dans ce cadre sont déterminées en référence à un taux historique et sont affectées d'un coefficient de minoration conduisant à ne compenser en réalité que 7 des moindres recettes. Ainsi, pour 502,5 millions d'euros de produit de taxe foncière non recouvré en 2018 en raison de l'exonération, seuls 17 millions d'euros ont été compensés aux communes en 2019. Dans ce contexte, il est nécessaire d'apporter une réponse aux inquiétudes des élus locaux quant au retour financier, même minimal, qu'ils peuvent espérer constater au bénéfice de leur collectivité locale, en incitant, en soutenant, en autorisant et en accompagnant la construction de logements sociaux. À cet effet, le présent amendement vise à transformer, à compter de 2022, le dispositif d'exonération de taxe foncière sur les constructions neuves de logements sociaux en dégrèvement, afin d'assurer une pleine prise en charge par l'État. Quel est l'avis de la commission

le Sénat en général, est favorable à l'adoption d'amendements de ce type, souvent déposés par notre collègue Philippe Dallier, visant à compenser au juste niveau le coût des exonérations de taxe foncière sur les constructions neuves de logements sociaux.

constructions de moins à la fin de l'année, sur un objectif de 500 000 logements. Nous sommes très en retard sur le logement social. On a abandonné la taxe d'habitation, qui assurait le lien entre l'habitant, l'usager des services de la commune

que vous n'aviez pas mesurées. Ce sera le boulet fiscal de votre mandature.

taxe d'habitation, avec les conséquences que les uns et les autres ont rappelées. Monsieur le ministre, les chiffres du logement social ne seront pas bons en 2020. Nous l'avons

se produira une grave crise du logement social et du logement intermédiaire et nous saurons, les uns et les autres, à qui et à quoi nous la devrons

Le débat sur le principe de la suppression de la taxe d'habitation a eu lieu à plusieurs reprises ; je ne l'ouvre pas à nouveau, mais je voudrais apporter quelques précisions, après ce que j'ai entendu. Tout d'abord, en 2023, quand la totalité de la taxe d'habitation sur les résidences principales- nous ne parlons que de celles-ci

que le système de compensation que nous avons mis en place, qui s'est traduit sur les douzièmes, permet une compensation à l'euro près ; il n'y a pas eu d'étranglement des collectivités. des départements ? De la même manière : la compensation se fait à l'euro près. Vous pouvez en contester les modalités, mais tel est bien le cas, je vous l'assure. Je vous invite à consulter les douzièmes pour voir ce qu'il en.

Cet amendement, proposé par ma collègue Sylviane Noël, vise à modifier l'article 1407 du code général des impôts, qui donne la possibilité aux communes dans lesquelles s'applique la taxe sur les logements vacants de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 5 % à 60 afin de lutter contre la pression immobilière. Seules les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants avec un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements peuvent actuellement utiliser ce levier fiscal.

Cet amendement tend donc à étendre la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires aux communes classées « station de tourisme », afin de maintenir les populations dans les stations et de permettre à ces territoires de contribuer à un développement touristique durable.

et elle apporte une première réponse à un sujet qui est de plus en plus prégnant sur les territoires touristiques, particulièrement dans les zones de montagne : les habitants,

à autoriser les aux collectivités locales qui le souhaitent à majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dans une proportion allant de 5 % à 100 %, et non plus à 60 % comme la loi l'autorise actuellement. Cette disposition permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu, notamment dans les zones urbaines denses classées A et A , d'avoir la possibilité de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d'habitation sur les résidences secondaires jusqu'à 100 %.

les taux restant inchangés pour les zones B et C. La demande en logements est particulièrement forte dans certaines zones. L'adoption de cet amendement permettrait donc de remédier en partie à ce problème.

résidents français contraints de résider dans un autre lieu en France pour des raisons professionnelles. Nous opérons le parallélisme des formes et nous ne voulons pas

les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l'instar des structures de statut public assumant les mêmes missions, selon les mêmes modalités de financement de leurs charges.

ainsi libellé : La parole est à Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous proposons de compléter la contribution économique territoriale (CET) par la création d'une taxe sur les actifs financiers des entreprises assujetties. La réforme de la taxe professionnelle a réduit l'indépendance et l'autonomie de gestion des collectivités territoriales.

de leurs recettes. L'imposition économique ne représente plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017, contre 482 euros pour la seule taxe Ce déséquilibre résulte d'un ensemble de dégrèvements, d'exonérations, de niches, de compensations en faveur des entreprises. Le champ d'action de la fiscalité locale étant réduit, les élus locaux se retrouvent contraints d'augmenter les impôts pesant sur les citoyens ou de restreindre leur offre de service public. Les dépenses d'action sociale ou de soutien à la vie culturelle et associative sont les premières concernées. Nous proposons de modifier la base de la CET afin qu'elle prenne en compte la réalité économique et les choix de construction capitalistique des entreprises, comme la suraccumulation du capital financier. ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Cela permettra, d'une part, d'abonder les ressources des collectivités, d'autre part, de contribuer à modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l'emploi et de l'investissement productif. Quel

qui souhaitent transformer leurs chambres en bureaux équipés et adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs. Vous connaissez l'état de la filière de l'hôtellerie,

serait de nature à réduire l'effet de ciseau entre l'évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en cette période de crise.

Cela reviendrait à nier l'autonomie de gestion des collectivités, ce qui ne nous semblerait pas opportun. La mesure proposée s'inscrit par ailleurs dans un contexte de réforme de la fiscalité locale et de perte par les départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti.

relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire rend obligatoire la mise en place de la collecte à la source de biodéchets d'ici à 2023. Pour cela, les collectivités territoriales peuvent mobiliser la fiscalité environnementale en instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative. La tarification incitative en matière de déchets permet la réduction de 20 % à 50 % de la production d'ordures ménagères et de meilleures performances du tri. Elle responsabilise l'usager en l'encourageant à adopter

pour le remboursement aux communes tient compte non seulement du dénominateur, mais aussi d'une forme de captation de recettes pour financer le prélèvement sur recettes qui sert de contribution de la France à l'Union européenne. Historiquement, dans les débats

Notre pays connaît un important déficit de logements sociaux, et la crise économique et sociale induite par l'épidémie de covid-19 entraînera un besoin croissant de logements abordables pour nos concitoyens. Il paraît donc pertinent de récompenser les communes rurales qui prennent leur part de la solidarité nationale en produisant de tels logements. Par ailleurs, comme le Gouvernement souhaite que les collectivités jouent un rôle central dans la relance de notre économie, une telle mesure peut être de nature à inciter les maires à produire du logement social, ne serait-ce que pour maintenir leur taux.

En l'état actuel, la clé de répartition n'est toujours pas satisfaisante. Aujourd'hui, nombre de collectivités rurales font un effort de solidarité au bénéfice de collectivités très peuplées,

du coefficient logarithmique de répartition. Il s'agit d'inciter le Gouvernement à réviser sa méthode de calcul au bénéfice des collectivités les moins bien loties, en faisant varier le coefficient non pas de 1 à 2, mais de 1 à 1,5. Quel

à Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à augmenter le taux du versement mobilité instauré en 2020 à Paris et dans les Hauts-de-Seine. En 2020, le versement aux 258 autorités organisatrices de la mobilité (AOM) aurait dû représenter plus de 9,4 milliards d'euros, pour moitié en province et en Île-de-France. Or la crise sanitaire est passée par là et les ressources du versement mobilité ont diminué proportionnellement aux baisses de revenus d'activité des entreprises de plus de onze salariés. Les AOM sont confrontées à une diminution de 10 % de leurs recettes au titre du versement mobilité, en plus de la baisse de 30 % des recettes tarifaires.

Ces baisses de recettes sont à mettre en balance avec la hausse des dépenses de nettoyage, de désinfection des véhicules et stations, d'installation d'une signalétique spéciale et d'achat de masques. La situation financière est grave, et le Gouvernement y répond en créant de la dette, le mécanisme des avances remboursables.

nous restaurerions une véritable contribution au service public de transports. Les entreprises qui souhaiteraient en être exemptées prendraient intégralement en charge le coût des transports de leurs salariés, comme cela est prévu. Aujourd'hui, le taux est le même, alors

Vous comprenez la logique : si les entreprises désirent tant surpayer leurs locaux professionnels, qu'elles assument une fraction équivalente des investissements en matière de transports. Il s'agit donc d'une mesure d'équité territoriale permet de restaurer l'attractivité à l'implantation d'entreprises, notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Quel

mais celle-ci est devenue obligatoire depuis, et les recettes sont intégrées dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale. Une telle situation peut créer d'importantes complications sur le terrain. Les syndicats dont les collectivités membres prélèvent la REOM

Lorsque la redevance est attaquée en justice, c'est à la communauté de communes émettrice du titre d'assurer la défense d'une redevance calculée par le syndicat. Cela suppose donc des échanges permanents entre le syndicat, qui assure la collecte, et la trésorerie des collectivités, qui prélève la redevance sans toujours disposer des moyens humains pour en assurer le suivi. Cette lourdeur administrative est encore plus difficile à gérer lorsque les collectivités concernées mettent en place la tarification incitative en vue de réduire les déchets sur leur territoire, car cela complexifie le calcul de la redevance et les relations avec les habitants. Cette situation nuit au développement de la tarification incitative, qui est pourtant un outil essentiel pour réduire les déchets résiduels. Pour simplifier la mise en oeuvre Pour simplifier la mise en oeuvre de la redevance et favoriser cette tarification incitative sans pénaliser les collectivités qui bénéficient d'une dotation majorée en intégrant la fiscalité déchets dans leur coefficient d'intégration fiscale, cet amendement vise à autoriser les collectivités à intégrer ces recettes dans leur coefficient d'intégration fiscale, y compris si c'est le syndicat auquel elles ont transféré la compétence qui prélève la taxe ou la redevance. Cette mesure sera sans répercussion sur le niveau de prélèvements, mais permettra aux collectivités qui ont transféré la compétence collecte de transférer également la gestion de la taxe d'enlèvement des

qui est de mesurer le degré d'intégration financière d'un EPCI à fiscalité propre en rapportant les produits fiscaux qu'il perçoit lui-même à l'ensemble des produits fiscaux du territoire. À droit constant, la mesure que vous proposez instituerait une rupture d'égalité entre les EPCI, en favorisant ceux qui ont transféré la gestion des déchets à un syndicat par rapport à ceux qui ont laissé cette compétence aux communes. C'est la raison pour laquelle

Ce n'est pas le cas pour les organismes privés non lucratifs assumant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires, ce qui méconnaît sans doute le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, avec un impact direct sur le reste à charge pesant sur les usagers, patients et résidents du secteur privé non lucratif. De ce point de vue, la réforme engagée de la taxe foncière dans le cadre de l'article 146 de la loi de finances pour 2020 doit permettre au législateur d'apprécier l'impact sur les finances sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives d'une évolution potentielle des taxes foncières, dans un contexte où il y a lieu d'attirer l'attention du ministère de l'économie et des finances sur la réalité de terrain, à savoir que la très grande majorité des baux civils ou professionnels conclus pour les locaux affectés à des activités sanitaires, sociales et médico-sociales prévoient explicitement l'imputation de la charge de la taxe foncière au locataire. L'hypothèse selon laquelle seuls les heureux propriétaires assumeraient en contrepartie de leur patrimoine la charge de la taxe et son éventuelle actualisation est donc totalement infondée s'agissant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.

les accompagnent. Nous voulons aussi saisir l'opportunité de fonder sur une connaissance objective les adaptations nécessaires des modalités d'évaluation, de neutralisation- à l'image de ce qui est prévu pour les monuments historiques -ou encore d'exonération- à l'image de ce qui est prévu pour les structures d'hospitalisation dédiées aux mutilés de guerre, dont une association de mutilés de guerre est propriétaire des locaux.

! Ce n'est pas assez cher ! L'article 196 de la loi de finances initiale pour 2020 prétendait « clarifier l'intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active

ne peut fonctionner à enveloppe constante. Pour cette raison, l'actuel projet de loi de finances prévoit une neutralisation du dispositif de garantie. Cependant, au regard des difficultés financières à venir des départements, dont nous avons amplement parlé, nous souhaitons qu'un rapport estimant la perte de produit de CVAE pour 2021 soit réalisé d'ici à la fin du premier trimestre afin de pouvoir anticiper l'éventuelle réactivation du mécanisme de garantie.

d'autre part, il nous reviendra d'examiner l'opportunité de refaire fonctionner le mécanisme de garantie en 2022 lors du prochain projet de loi de finances, lorsque nous aurons tiré quelques enseignements de la situation passée. l'année 2021, c'est à l'État, et non à la péréquation horizontale, d'assurer la compensation des pertes. Je rappelle que nous avons voté, sur l'initiative de la commission, un amendement en ce sens en première partie.

pour y souscrire et par les types d'activités retenus, il est proposé que les personnes et organismes redevables de la CFE bénéficient, au titre des cotisations dues au 1 janvier 2020 et au 1 janvier 2021, d'une franchise de 3 000 euros.

ont eu des conséquences économiques majeures sur le tissu économique de notre pays. S'il serait malhonnête de minimiser l'importance des mesures de compensation et de soutien apportées par le Gouvernement,

de réduire le montant de la CFE pour l'année 2021, au prorata de la période de fermeture des établissements. Les décisions de fermetures administratives ayant été décidées par l'État, le manque à gagner fiscal pour les communes et EPCI à fiscalité propre serait compensé par une majoration de la DGF. Quel est l'avis

général. L'article 42 du projet de loi de finances prévoit de supprimer la taxe sur les services funéraires.